J'appelle en discussion les articles 77 à 78 et les amendements portant articles additionnels, qui sont rattachéspour leur examen aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

en automatisant le rééquilibrage et en prévoyant déjà le taux de minoration, afin d'alléger le plus rapidement possible la pression fiscale pesant sur ces communes. Les communes ne doivent plus être obligées de payer le FNGIR, alors qu'elles ne touchent plus aucune dotation par ailleurs. Il s'agit d'un amendement de bon sens. Déjà déposé l'année dernière, il reste d'actualité. Il avait été indiqué à M. Courtial que l'adoption du présent dispositif aboutirait concrètement à faire financer les minorations du FNGIR par les autres collectivités.

traduit une préoccupation légitime, qui a déjà été exprimée, concernant les dysfonctionnements avérés du dispositif. Toutefois, l'adoption de cet amendement aurait pour effet de minorer le reversement aux collectivités bénéficiaires et ferait donc un grand nombre de perdants

c'est pour vous faire partager ma satisfaction, mes chers collègues, de voir enfin un changement profond dans l'approche gouvernementale du traitement de l'outre-mer dans la répartition des dotations. Très explicite à cet égard est le document d'évaluation du PLF pour l'article 78, qui constate que la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, la Dacom, en dépit de son mode de calcul, se révèle moins favorable au total que ce que pourrait amener l'application des règles de péréquation applicables en métropole. Tout y est dit ! Cela peut paraître anodin aux yeux de certains, mais, pour les Ultramarins, et pour moi tout particulièrement, c'est une avancée considérable. Depuis mon élection en 2008, je n'ai eu de cesse au sein de cette assemblée de dénoncer le traitement inique des outre-mer et de présenter des amendements pour mettre fin à cette situation. En vain ! La Cour des comptes a fini par le reconnaître en 2017. Le Président de la République l'a admis durant la réunion organisée à l'Élysée avec les élus locaux d'outre-mer, lors du grand débat, et le Gouvernement concrétise aujourd'hui les engagements pris. Rendez-vous compte, cela faisait des années que les plus pauvres des territoires de la République ne percevaient pas ce à quoi ils avaient droit, subissant même une double peine avec la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) qui les a lourdement pénalisés, contrairement aux communes les plus fragiles de l'Hexagone. Certes, nous ne pouvons pas tout remettre à plat d'un seul coup. La proposition du Gouvernement d'une mise à niveau sur cinq ans, avec la création d'une dotation de péréquation des outre-mer, dotée de 18,3 millions d'euros supplémentaires tous les ans, jusqu'à atteindre 91 millions d'euros, montant estimé de l'écart entre les communes des DROM et celles de l'Hexagone, est à saluer. Néanmoins, pour parvenir à un réel ajustement à une réelle mise à niveau, des mesures exceptionnelles doivent être envisagées, notamment pour financer des plans d'accompagnement pour les communes les plus en difficulté et pour lesquelles la Cour des comptes reconnaît que, « malgré un train de vie très rigoureux, le retour à l'équilibre n'est pas envisageable par les seuls moyens de la commune. Enfin, je veux terminer sur ce qui, à mon avis, est une des causes du refus de voir depuis de si nombreuses années la réalité du traitement injuste des collectivités d'outre-mer dans la répartition des dotations : leurs faibles poids et représentativité au sein du Comité des finances locales (CFL), instance qui a la haute main sur les dotations. Que pèsent 212 communes ultramarines face à près de 36 000 dans l'Hexagone ? Comment garantir dans ces conditions une réelle prise en compte des enjeux ultramarins au sein du CFL, hors gestion de crise ? Jusqu'à quel point êtes-vous prêts à faire jouer la solidarité nationale pour les outre-mer ? Telle est en fait la question.

crainte avait, dans un premier temps, été levée, puisque le Gouvernement avait accordé une garantie, sans limites de temps, en matière de DSR, aux communes ayant fusionné avant le 1 janvier 2018. le présent article supprime cette disposition à compter de 2023. Pour nombre de communes connaissant une croissance démographique exponentielle, le seuil des 10 000 habitants sera dépassé en 2023. L'exemple de la commune de Fillière, en Haute-Savoie, est flagrant. Avec cette disposition, elle perdra 150 000 euros en 2023, soit 50 % du montant de la DSR, en vertu d'une garantie de sortie, puis 300 000 euros dès 2024. Pour cette commune, comme il en existe bien d'autres, la dotation ne pourra être compensée par le bénéfice de la dotation de solidarité urbaine, car cette dotation est distribuée en fonction d'un indice synthétique prenant en compte le potentiel fiscal par habitant, le poids des logements sociaux, le poids des bénéficiaires des allocations pour le logement et le revenu par habitant. Cette perte, conjuguée à la perte du bonus de la dotation globale de fonctionnement, ou DGF, réduira considérablement la capacité d'investissement de bon nombre de communes. Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition, afin de garantir aux communes nouvelles créées avant le 1 janvier 2018, et dont la population ne cesse d'augmenter,

de leur création « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux ». Le Gouvernement semble d'avis que ces dispositions doivent s'appliquer à toutes les communes nouvelles remplissant les conditions d'éligibilité, indépendamment de leur mode de création. L'adoption de cet amendement clarifierait

L'article 78 du PLF pour 2020 propose de conditionner la perception de cette dotation de compensation aux seules communes-communautés, issues du 2 août 2019, regroupant moins de 150 000 habitants et n'adhérant pas à un autre EPCI à fiscalité propre. Une commune-communauté, qui a vocation à reprendre des compétences anciennement intercommunales, ne peut se voir supprimer

de la loi, qui facilite le regroupement de communes-communautés, et que nous avons votée en août 2019. Le présent amendement vise à rétablir le principe de la perception de l'ancienne dotation de compensation de l'EPCI, supprimée, pour l'ensemble des communes-communautés qui souhaiteraient en disposer.

en tout état de cause, dans la mesure où les communes-communautés sont considérées, au regard la DGF, et en particulier de la dotation de compensation de la part salaires, comme des communes isolées. Elles la perçoivent déjà.

visibilité. Nous revenons à un régime de droit commun pour toutes les communes nouvelles, en mettant en effet un terme au bénéfice de la DSR à vie

Ces communes ont d'ores et déjà bénéficié de dispositions avantageuses par rapport aux autres communes, pendant de nombreuses années. Il convient de ne pas accentuer cette dérogation. Je demande donc le retrait

le rappelle, le pacte de stabilité des nouvelles communes repose sur des principes clairs : la protection des communes contre la baisse des dotations pendant leurs premières années d'existence et une bonification des dotations-

Le PLF pour 2020 réaffirme ces principes, qui étaient parfaitement connus des communes au moment où elles ont choisi de fusionner.

En outre, cher collègue Sido, vous affirmez qu'il ne faudrait pas donner aux communes nouvelles une incitation financière, une sorte de carotte, mais, dans ce cas, pourquoi a-t-on instauré un coefficient d'intégration fiscale pour encourager à

Eh bien, je suis désolé, mais il y a eu une période transitoire et elle est terminée. Il faut considérer les communes nouvelles comme des communes, sans quoi les choses ne sont pas claires

qu'elles deviendront une seule et unique commune ; c'est un choix. Eh oui ! Il faut dire les choses comme elles sont ; sinon, on est dans l'ambiguïté la plus totale. La parole est à M. Philippe

Les communes nouvelles sont nées d'un mouvement des élus, qui voulaient se regrouper pour mettre en commun un certain nombre de services. Il y a certes eu des incitations, mais la fusion a gardé son

l'amendement n° II-429 rectifié. Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du FPIC. Ces prélèvements fragilisent leur situation budgétaire en diminuant leurs capacités d'investissement, pourtant indispensables pour maintenir une offre touristique de qualité et renforcer leur attractivité, ce qui génère des recettes

Afin de mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les communes touristiques, la loi de finances pour 2019 a porté la majoration de la population totale de 1 à 1,5 habitant par résidence secondaire située dans les communes de moins de 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %. Toutefois, la condition relative au potentiel fiscal pénalise fortement les communes touristiques, qui, en raison de leur activité, peuvent bénéficier de recettes fiscales supérieures à la moyenne des communes de même strate, mais sont également soumises à des charges touristiques bien plus élevées. Leurs dépenses d'entretien sont, en effet, plus importantes, en raison de l'accueil de la population touristique et du dimensionnement de leurs équipements de loisirs et de l'ensemble de leurs réseaux routiers ou d'assainissement, par exemple. Le rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2019 confirme les disparités des dépenses par habitant selon la taille et les caractéristiques économiques et géographiques des collectivités, indiquant que, « en dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes.

afin de mieux prendre en compte leurs charges spécifiques, à condition que leur potentiel fiscal ne soit pas trop élevé. Au total, 1 189 communes touristiques ont pu en bénéficier.

M. Didier Marie. Cet amendement, adopté par le Sénat l'an dernier, vise à éviter que les collectivités les moins riches supportent, à la place des collectivités les plus riches, le financement de la péréquation verticale. En effet, chaque année, la dotation forfaitaire des communes est écrêtée pour financer des « contraintes internes » à la répartition de la DGF, en particulier la progression des dotations de péréquation- DSU et DSR. Afin de ne pas faire supporter la charge de cette minoration sur les communes les moins favorisées, qui ont vocation à bénéficier pleinement de la hausse des dotations de péréquation, la loi prévoit que l'écrêtement est réalisé sur la dotation forfaitaire des communes qui présentent un certain niveau de potentiel fiscal par habitant. Ce sont ainsi les communes avec les dotations forfaitaires les plus élevées qui financent la progression de la péréquation pour les communes les plus en difficulté. Toutefois, la contribution au redressement des finances publiques a minoré la dotation forfaitaire des communes. Elle a même fait disparaître la dotation de certaines d'entre elles. Ces communes, pour lesquelles la DGF est négative, échappent au financement de la progression des dotations de péréquation, alors même qu'elles peuvent présenter un niveau de richesse très élevé, lequel se traduit par un potentiel fiscal par habitant qui est jusqu'à quinze fois supérieur au seuil d'écrêtement.

Cette évolution permettrait d'assurer une plus grande solidarité entre les collectivités et de mieux répartir la charge entre les communes écrêtées. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

on constate qu'un certain nombre de communes riches, qui, certes, ne perçoivent plus DGF, et pour cause, ne contribuent pas à la solidarité entre nos territoires. Cette situation est dommageable. Même si j'entends la remarque de M. le rapporteur spécial

ces dotations avaient connu une progression inédite entre 2015 et 2017, puisqu'elles avaient progressé de 180 millions d'euros chacune.

dans une logique de péréquation et au regard d'indicateurs adaptés aux spécificités de l'outre-mer. Afin de renforcer cette logique, le présent amendement tend à accroître l'enveloppe dédiée à la partie péréquée de la nouvelle dotation d'aménagement des communes et Néanmoins, le dispositif prévoit un mécanisme de garantie pour qu'aucune commune ne voie son attribution par habitant diminuer au final. Ainsi, le total par habitant des deux dotations ne pourra pas régresser. Compte tenu de la hausse globale de l'enveloppe, toutes les communes connaîtront une augmentation par habitant de leur dotation de péréquation. à ajouter trois critères dans le calcul de la dotation de péréquation, en plus du potentiel financier et du revenu, de manière à mieux retranscrire les spécificités et besoins des communes d'outre-mer : le nombre d'enfants, le nombre de bénéficiaires du RSA et le nombre de bénéficiaires des aides au logement. Enfin, il tend à prévoir une meilleure prise en compte des charges de centralité supportées par les « villes capitales » des départements d'outre-mer, en majorant la dotation qui sera versée aux chefs-lieux de département et d'arrondissement comptant plus de 10 000 habitants. Ces critères complètent les deux critères déjà proposés dans l'article, à savoir le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant.

financée par « de l'argent frais », c'est-à-dire par une augmentation de la DGF de 15 millions d'euros. Cette dotation d'intercommunalité a montré son intérêt. Il serait opportun que le Gouvernement participe à cette augmentation de la péréquation.

pour le calcul de la dotation d'intercommunalité que nous n'avons pas réussi à faire financer par l'État à l'instant. Les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le CIF est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle de l'année précédente. De même, les communautés de communes dont le CIF est supérieur à 0,5 perçoivent aussi une dotation par habitant au moins égale à celle de l'année précédente. Cela étant, l'écart entre les deux

L'adoption de cet amendement changerait l'équilibre de cette dotation, puisque cette garantie complémentaire pour certaines communautés de communes se traduirait par une moindre attribution pour les EPCI ne bénéficiant pas de la garantie.

d'accord. Il s'agit de faciliter la procédure de reversement et d'inciter les collectivités à recourir au dispositif. Si un conseil municipal ne délibère pas sur la proposition de l'EPCI, il sera donc réputé l'avoir acceptée.

de l'exercice des compétences, la neutralité financière doit être garantie. En l'état du droit, de telles restitutions de compétences, parce qu'elles entraînent également des restitutions de produits fiscaux, se traduisent par une baisse du coefficient d'intégration fiscale de l'établissement, donc par une diminution de la dotation d'intercommunalité, sans que les communes perçoivent pour autant un surplus de dotations. Les règles de répartition des concours financiers de l'État favorisent donc l'exercice des compétences au niveau intercommunal plutôt que communal, sans aucune justification évidente. Nous l'avions souligné lors des débats sur le projet de loi Engagement et proximité, peut-être l'intercommunalité est-elle allée trop loin en matière d'intégration fiscale. Dans un contexte financier difficile, ces règles empêchent ou dissuadent les élus de faire prévaloir le principe de subsidiarité dans la répartition des compétences locales. Cet amendement tend que le coefficient d'intégration fiscale d'un EPCI à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de sa dotation d'intercommunalité ne pourra, à l'avenir, être inférieur à son niveau de 2019, de 2019, et que les EPCI à fiscalité propre qui bénéficieront de cette garantie devront en reverser le produit à leurs communes membres au prorata de leur population, sous la forme d'une dotation de territorialisation qui contribuera au financement des compétences restituées aux communes.

Engagement et proximité. Dans le cadre de la nouvelle carte intercommunale, certains EPCI devront rendre des compétences à leurs communes membres, ce qui se traduira par une diminution de leur coefficient d'intégration fiscale

de cet amendement introduisent une sorte de flux de la dotation intercommunale vers les communes. La dotation d'intercommunalité repose sur le principe du coefficient d'intégration fiscale,

La dotation d'intercommunalité en tient logiquement compte : elle augmente au fur et à mesure de l'augmentation du CIF, ce qui est tout à fait logique.

un EPCI dont le CIF diminue et qui exerce donc moins de compétences voit sa dotation baisser. Dans une enveloppe fermée, les sommes dégagées par cette baisse viennent abonder la dotation des EPCI qui s'intègrent. C'est le principe même de la dotation, réaffirmé par le législateur lors de la réforme votée en loi de finances pour Ce sont donc bien les EPCI dont l'intégration augmente ou reste stable

pour ceux qui sont en voie de désintégration. C'est incompréhensible, infondé et inutile.

que le Sénat s'attache à relever dans la période actuelle ? Cet enjeu peut se résumer d'un mot : proximité. Il fut un temps où nous avons voulu forcer l'extension des périmètres des communautés de communes et, concomitamment, et, concomitamment, leur intégration. Ce temps est révolu. Ce qui a été fait est fait. La réalité d'aujourd'hui est différente de celle de l'époque où ces instruments ont été conçus.

par l'amoindrissement de l'intégration de certaines autres communautés de communes ? Non, bien évidemment : le système ne fonctionne pas pour permettre de s'intégrer davantage avec l'argent de ceux qui s'intégreront moins.

effet, si on laisse jouer le mécanisme du coefficient d'intégration fiscale, les gagnants sont ceux qui arrivent à une intégration de 100 %, en vidant financièrement les communes. Personne ne veut cela, cet instrument est devenu fou ! C'est la raison pour laquelle, après bien des interventions, les

occupés à vendre à leurs élus les montages les plus ingénieux - je m'exprime de manière positive -, pour essayer de prélever quelques centaines de milliers d'euros de dotations à leurs voisins, en jouant sur un coefficient d'intégration qui est en partie «

financièrement les communautés qui adopteraient cette souplesse, au profit de celles qui font la course au CIF, en intégrant toujours plus

prévoir des dispositions, appelées exceptions, pour adapter les mécanismes financiers à l'évolution du monde. Si nous ne conduisons pas une réforme véritable et profonde des dotations aux collectivités, nous n'en sortirons jamais

Elle est arrivée à maturité. Aujourd'hui, il s'agit non plus de forcer à l'intégration maximale, mais de trouver, comme cela a été dit, le meilleur arrangement possible pour rendre le meilleur service aux habitants,

Notre collègue Alain Richard évoquait ces directeurs financiers qui arrivent avec des statistiques et des tableaux de bord, pour expliquer que l'intégration financière doit se poursuivre. Cela a créé dans de nombreuses intercommunalités un renforcement de la superstructure intercommunale, au travers de

Le scrutin est ouvert.

n° II-27. Compte tenu de l'amendement n° I-73 adopté par la commission des finances à l'article 5 du présent projet de loi de finances, qui vise le rapport vise le rapport que le Gouvernement aura à remettre au Parlement sur les conséquences financières de la réforme du financement des collectivités territoriales proposée, cet amendement tend à supprimer les dispositions introduites à l'Assemblée nationale, qui demandent un rapport sur le même sujet, mais dans un calendrier différent.

Le Gouvernement souhaite bien sûr maintenir le calendrier de la réforme fiscale proposée en PLF et adoptée par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une entrée en vigueur en 2021. Dans ces conditions, rien ne justifie la suppression du rapport demandé par les députés pour juillet 2020. Le calendrier proposé par l'Assemblée nationale est en outre parfaitement synchronisé avec les travaux qui seront menés par le Comité des finances locales au premier semestre 2020. Le Gouvernement est donc défavorable

d'abord, elle reflète imparfaitement les différentes strates de collectivités, puisque la carte a considérablement évolué entre 2011 et 2020. Il conviendrait donc de revoir la pondération entre les différents niveaux, notamment entre les communes et les EPCI. Par

Par souci de continuité, la nouvelle dotation de biodiversité qui absorbe l'actuelle dotation Natura 2000 doit être inscrite sur le même programme.

avec les délais de publication propres à la DGF. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire la dotation de biodiversité sur les crédits de

répartis de la façon suivante : 55 % pour les sites Natura 2000, 40 % pour les coeurs de parcs nationaux et 5 % pour les parcs marins.

Par ailleurs, les moyens consacrés à la part Natura 2000 ont été calibrés de manière à permettre aux communes qui étaient déjà éligibles à la dotation en 2019 de ne pas perdre de ressources, alors même que le nombre de communes concernées par un site Natura 2000 est en augmentation, comme l'est le nombre de communes éligibles à la dotation, du fait d'un desserrement du critère de potentiel fiscal.

Il s'agit d'abaisser le seuil de population applicable aux communes bénéficiaires du dispositif Natura 2000 de 10 000 à 5 000 habitants, et ce afin de permettre aux collectivités concernées de disposer d'une dotation plus importante. Je rappelle que, en 2019, 1 118 communes se sont réparti les 5 millions d'euros de la nouvelle dotation Natura 2000. Si l'effort financier consacré au verdissement de la DGF est un signe important pour les territoires, il représente en moyenne moins de 5 000 euros par commune. Le détail de la répartition fait apparaître que près de la moitié des 1 118 communes bénéficiaires classées en zone de montagne. Cela peut sembler cohérent au regard de l'objectif du réseau Natura 2000, qui est un outil de préservation de la biodiversité et de prise en compte des enjeux afférents dans les activités humaines. Pour autant, les communes de montagne ne bénéficient que d'une part assez faible des 5 millions d'euros car celle-ci est calculée en fonction du nombre d'habitants et de la proportion du territoire de la commune couvert par un site Natura 2000. Ainsi, certaines communes classées en zone de montagne touchent moins de 200 euros. Pourtant, Pourtant, ainsi que le souligne le dernier rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales, « à population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont [ ...] plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour les autres communes. En dessous de 10 000 habitants, c'est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Plus les communes sont grandes, plus les différences s'estompent

en matière de dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité. L'Assemblée nationale, pour tenir compte de la création d'un onzième parc cette année,

intervenu en 2017. Cet amendement vise donc à faire en sorte qu'en 2020 près de 174 ensembles intercommunaux et 5 779 communes puissent bénéficier d'une garantie pérenne de sortie progressive de l'éligibilité au reversement du FPIC, et ce sur quatre années. Quel est l'avis de la commission ? Cet

Il s'agit aussi parfois de territoires industrialisés ou anciennement industrialisés bénéficiant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), qui, depuis la mise en oeuvre de cette réforme, se trouve incorporée au potentiel fiscal, alors que les autres bases de calcul de celui-ci ne témoignent pas d'une richesse évidente. Il s'agit non pas de remettre en cause ce principe de péréquation, mais de limiter les impacts excessifs qu'il a sur certains territoires dont les critères d'appréciation de la richesse sont à des niveaux assez modestes. Dans l'attente d'une réforme plus structurelle, il convient de minorer

résoudre la question du traitement donné à une dotation de compensation justifiée par une réforme très lointaine, alors que la situation des communes auxquelles elle est accordée

pour le calcul de la DGF dans les communes touristiques. La population prise en compte pour le calcul de la DGF résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée de 1,5 habitant par résidence secondaire. Cette majoration ne prend pas suffisamment en compte, d'une part, la diversité des modes d'hébergement dans les communes touristiques, d'autre part, l'augmentation du nombre de résidences secondaires ces dernières années. territoriales, publiée au mois de janvier 2017, souligne que les dépenses de fonctionnement par habitant sont en moyenne plus élevées pour les communes touristiques. Parmi les communes touristiques, les communes de montagne ont des dépenses par habitant très supérieures. Quel

Ces prélèvements fragilisent leur situation budgétaire en diminuant leurs capacités d'investissement, pourtant indispensables pour maintenir une offre touristique de qualité et renforcer leur attractivité, qui génère des recettes de TVA pour l'État et crée des emplois. Face au changement climatique, les petites communes touristiques devraient pouvoir conserver des moyens d'investir afin de préserver leur vitalité économique, sociale et territoriale

L'autre jour, on m'a fait savoir à grands cris que la République était une et indivisible. Vous avez la preuve que c'est faux

Toujours sur la base de ce critère, il est apparu que le solde des montants reversés et perçus par les ensembles intercommunaux d'outre-mer diminuerait très légèrement. En d'autres termes, l'application des règles de droit commun en matière de FPIC pourrait modifier la répartition des contributions et versements entre les ensembles intercommunaux en outre-mer, mais n'aurait pas d'impact sur les territoires métropolitains.

En effet, à enveloppe constante du FPIC, l'adoption de cet amendement conduirait à transférer 30 millions d'euros des ensembles intercommunaux métropolitains vers les ensembles intercommunaux ultramarins. En outre, rien ne semble justifier que l'octroi de mer soit comptabilisé comme une ressource pour le calcul de la DGF, mais pas pour le FPIC. Procéder ainsi serait assez curieux.

et travaillons avec l'ensemble des groupes pour tenter de trouver la moins mauvaise solution possible, car il y a là manifestement un problème. Enfin, vous avez évoqué le statut de l'octroi de mer.

je suis tout à fait conscient de la nécessité de cette péréquation : Paris doit participer à la solidarité, à la fois en Île-de-France et à l'échelon national.

qu'elle devait au regard des différents critères de répartition du FSRIF. Les conséquences ont été importantes. Nombre de communes n'ont pas bénéficié des autres modalités de plafonnement- à savoir 11 % des dépenses réelles de fonctionnement ou alors une variation de la contribution

à la solidarité. Ils pourront également mesurer l'évolution des dépenses de leur collectivité, en fonction de l'effort de solidarité auquel elles doivent se soumettre.

Les premiers retours des départements font globalement apparaître que les critères d'attribution de cette dotation ont été à géométrie variable. Son mode de calcul et de versement rend par ailleurs le rythme de perception beaucoup moins linéaire que ne l'était la DGE. Un grand nombre de départements se sentent perdants, sans qu'ils aient pu anticiper la situation. C'est pourquoi un premier bilan est indispensable afin d'ajuster et d'améliorer le fonctionnement de la

interdépartementale à travers la fusion des prélèvements opérés au titre des trois fonds de péréquation assis sur les droits de mutation à titre onéreux perçus par les conseils départementaux : le fonds national de péréquation

Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du RSA est transférée à l'État, des modalités de neutralisation financière sont prévues par l'article 25 du projet de loi de finances.

interdisent que le budget d'une commune membre prenne à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. En outre, à la différence des EPCI à fiscalité propre, les EPCI peuvent recourir aux contributions directes de leurs membres et les les moduler. Il me semble qu'une ouverture trop large des fonds de concours serait susceptible de remettre en cause les principes propres au transfert de compétences des communes vers un EPCI. J'ajoute qu'une telle extension serait un facteur d'endettement supplémentaire

Madame la ministre,

Ce critère exclut toutes les communes, pourtant éligibles à la DETR, qui appartiennent à un EPCI de plus de 75 000 habitants. Alors que les logiques de regroupement intercommunal à plus grande échelle ont été encouragées, la répartition de la DETR pénalise cet effort de rationalisation de la carte intercommunale. Il s'agit donc de faire correspondre effectivement la base de calcul de la DETR entre les départements avec les populations des communes éligibles à la DETR.

de la population des EPCI éligibles. Cet amendement tend à remplacer cette population par celle des communes éligibles. Toutefois, le Gouvernement, après un travail très poussé sur les variations annuelles des enveloppes départementales de DETR, a souhaité les stabiliser pour l'année prochaine, ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, afin de mener un travail

de l'ordre de 149 928 euros. Les opérations les plus coûteuses, bénéficiant de fortes subventions, absorbent une part importante de l'enveloppe de la DETR, même si les pratiques varient très fortement d'un département à l'autre. À titre de comparaison, le montant moyen des subventions attribuées à la demande des sénateurs au titre de feue la réserve parlementaire était de 6 788 euros en 2017, et le coût total moyen des projets subventionnés de 102 850 euros. Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes rurales pour boucler le financement de petits projets, cet amendement vise à réserver une part égale à 15 % de l'enveloppe départementale de DETR aux projets dont le coût n'excède pas 50 000 euros. Les subventions resteraient attribuées par le préfet de département.

Je serais heureux de me rallier à la philosophie de Mme la ministre, qui considère qu'il faut éviter de créer des rigidités supplémentaires dans l'attribution des subventions,

des écrans radars de la dotation d'équipement des territoires ruraux, dont la moyenne des attributions atteint un peu plus de 40 000 euros. Nous voudrions que

de s'emparer du dispositif pour pousser les dossiers des communes rurales avec lesquelles ils sont en contact. Nous considérons que la réforme s'est faite au détriment des communes rurales et que notre devoir est de rétablir le fléchage des crédits de l'État vers leurs investissements, qui sont trop souvent ignorés.

Nous savons que les conseils départementaux, bien avant la disparition de la réserve parlementaire, ont souvent créé des dispositifs très souples, très rapides, très réactifs et très agiles pour accompagner les petits investissements en milieu rural.

par le préfet de région. Hormis le cas où un seul département serait éligible à une attribution de subvention, il est prévu que la consultation des présidents de conseils départementaux de la région est un préalable aux décisions d'attribution.

de la commission ? Cet amendement tend à ce que le préfet de région attribue les subventions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements après avis des présidents de chaque conseil départemental. Nous y sommes défavorables, car ce dispositif nous semble comporter plusieurs risques. Cela conduirait à ce que les présidents des conseils départementaux donnent leur avis sur les projets de subventions de leurs voisins,

faible ampleur des petites communes ne sont plus du tout défendus, puisque seule la DETR peut y répondre.

soient principalement attribuées par le préfet de département, et non plus par le préfet de région. En pratique, les préfets de région délèguent cette tâche aux préfets de département, qui la subdélèguent parfois aux sous-préfets d'arrondissement, ce qui ralentit considérablement le circuit de décision.

Afin que les préfets de région puissent néanmoins opérer une forme de redistribution entre les départements, s'ils l'estiment nécessaire, et financer d'éventuels projets d'ampleur régionale, une quote-part égale à 20 % du montant de la DSIL est réservée, qui continuerait à être répartie par le préfet de région. En outre, cet amendement tend à créer une commission départementale des investissements locaux, chargée de contrôler la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la part départementale de la dotation de soutien à l'investissement local. Il

Cette commission, modelée sur l'actuelle commission DETR, mais disposant de compétences renforcées, traitera des deux dotations. Elle serait ainsi destinataire de la liste des demandes de subvention attribuées au préfet de département et appelée à formuler un avis sur la liste complète des subventions projetées.

alors que l'on nous a vendu la suppression de la réserve parlementaire comme une mesure de transparence. Il faut garantir aux maires, aux communes et à nos concitoyens

qui ont été signés pour quatre ans, en 2017, entre l'État et les EPCI ou les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux

l'un des deux premiers critères, mais qui seraient visées par le programme national de renouvellement urbain (PNRU). Par ailleurs, ce nouveau critère semble largement redondant par rapport à l'un des trois critères actuels.

sous la forme d'une majoration de leur taux de subvention. Cette faculté, ouverte par la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, est entièrement à la main des préfets qui en définissent eux-mêmes les modalités d'usage. Elle est source d'opacité et de déconnexion des dotations avec les besoins effectifs du terrain. À enveloppe constante, cette majoration du taux de subvention pour certaines collectivités revient surtout à diminuer les dotations des collectivités n'ayant pas voulu être intégrées au processus de contractualisation ou n'ayant pas pu respecter leur contrat pour accroître celles des collectivités ayant respecté ce contrat. Cette faculté revient donc à organiser le transfert de certaines collectivités, considérées comme insuffisamment maîtresses de leur gestion financière, vers d'autres collectivités jugées plus vertueuses sur le plan financier. Un tel transfert est d'autant plus paradoxal qu'il tend à nuire aux collectivités connaissant déjà des difficultés financières. Cet amendement a donc pour objet d'encadrer cette faculté. Le préfet de région ne pourrait en faire usage que lorsqu'il est constaté, en fin d'exécution, que l'ensemble des crédits n'ont pas été consommés. Préalablement à la décision de majoration du taux de subvention, il serait tenu de motiver sa décision dans un avis rendu à la commission DETR du département sur lequel est située la collectivité en question. Cet avis permettrait à la commission DETR d'être informée et de s'assurer qu'aucun autre projet ne verrait ces crédits mieux employés.

Je ne reviendrai pas sur le dispositif qui vient d'être présenté. Il nous semble que cette procédure ferait surtout peser un risque de sous-exécution des crédits en fin d'année, alors que le préfet a de toute façon la latitude d'accorder une majoration de DSIL.

d'un établissement public territorial de bassin ou d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau d'imputer les contributions versées pour financer des investissements dans le grand cycle de l'eau en section d'investissement, contrairement à la situation actuelle où elles sont imputées exclusivement aux dépenses de fonctionnement.

Le projet de loi Engagement et proximité a prévu la souscription par toutes les communes d'une assurance destinée à couvrir les coûts engendrés par l'octroi de la protection